La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix.

est à Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à dissocier, dans les délégations possibles de l'État à la métropole du Grand Paris (MGP), les compétences relatives aux aides au logement et celles relatives à l'hébergement. La métropole du Grand Paris exercera la compétence d'attribution d'aides financières au logement social à compter de l'adoption de son plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Cette prise de compétence doit marquer une nouvelle étape pour le développement du logement social dans l'agglomération parisienne et sa répartition géographique plus équilibrée. L'association de ces financements à la délégation des aides de l'État au logement pourrait constituer un effet levier important pour ce développement et faciliter les procédures d'attribution par le biais d'une instruction unifiée. Cependant, cette délégation à la métropole est actuellement indissociable de celle des compétences liées à l'hébergement. Historiquement et jusqu'à aujourd'hui encore, seules les aides à la pierre ont été déléguées aux collectivités franciliennes. est actuellement la seule collectivité du périmètre métropolitain titulaire de la délégation des aides au logement et elle l'exerce indépendamment des compétences liées à l'hébergement, qui demeurent de la responsabilité directe de l'État. La délégation de la compétence hébergement n'a jamais été mise en oeuvre en Île-de-France et nécessite, au vu des caractéristiques et de l'importance qu'elle revêt dans l'agglomération parisienne, une négociation spécifique et dissociée de la question du logement. L'impossibilité de dissocier ces compétences pourrait donc conduire à une impasse pour engager leur décentralisation. Nous constatons, en outre, que l'État n'a nullement l'obligation de déléguer ses compétences à la métropole, pas plus que la métropole n'a celle de les demander

compte tenu des enjeux immenses d'articulation entre le logement et l'hébergement sur un territoire, en particulier dans la métropole du Grand Paris. C'est la garantie d'une gestion cohérente de la politique de l'habitat, au sens large, avec pour objectif partagé de garantir un accès au logement pour tous. Logement et hébergement seront d'ailleurs traités comme un tout cohérent au travers du futur plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement de la MGP.

libellé : La parole est à M. Olivier Henno. L'objet du présent amendement est de compléter l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation afin que les organismes d'HLM soient associés de droit à l'élaboration des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT). Rappelons que ces opérations visent, notamment, à adapter et à moderniser le parc de logements afin de favoriser la mixité sociale. Les organismes d'HLM mènent très fréquemment des opérations immobilières ou d'aménagement qui concourent à la revitalisation des centres-villes. À titre d'illustration, ils sont particulièrement présents et contribuent fortement au déploiement sur le terrain du programme national Action coeur de ville, avec près de 90 % des 9 600 logements financés par Action Logement. Le succès des Le succès des ORT passe par la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux susceptibles de concourir à leur réalisation. Il est par conséquent indispensable que le représentant de ces organismes, lorsqu'il n'est pas signataire de la convention d'ORT, soit consulté sur son projet au cours de sa phase d'élaboration. Quel

. Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ÉLAN), les ORT permettent de mettre en oeuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l'immobilier de loisir. Un bilan de la mise en oeuvre des moyens, des outils et des méthodes mis à la disposition

Cela permettra ensuite d'engager un travail en vue d'une meilleure prise en compte des enjeux liés à ces territoires singuliers. La parole est à M. Pascal Martin, pour

trop contraignantes. L'article 47 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne autorise déjà les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des travailleurs saisonniers. Cependant, toutes les difficultés subsistantes, il faut actionner tous les leviers pour diversifier l'offre de logement à destination des travailleurs saisonniers. À ce titre, les organismes de foncier solidaire (OFS) peuvent jouer un rôle dans le développement de l'offre de logements pour les travailleurs saisonniers. C'est pourquoi il est proposé, par cet amendement, d'étendre à cette fin l'habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance.

Néanmoins, nous avions souhaité, dans le cadre de cette habilitation à légiférer par ordonnance, pouvoir ouvrir à titre subsidiaire- j'insiste sur cette précision importante -la possibilité d'utiliser les mécanismes des OFS et des BRS pour développer l'offre de logements intermédiaires et, dans un certain nombre de cas, de locaux d'activités.

l'objet des OFS à la rénovation des copropriétés, à leur permettre d'être tiers financeurs, et à adapter les conditions de majorité à réunir lorsque l'assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur ce contrat global de rénovation. La parole

si les bailleurs sociaux détiennent la qualité de maître d'ouvrage lors de la réalisation de logements à usage locatif aidés par l'État, le droit actuel ne précise pas si cela inclut les logements réalisés pour le compte d'un organisme de foncier solidaire dans le cadre d'un BRS. Cette situation provoque des incertitudes juridiques quant aux opérations imbriquant un équipement public au sein d'un ensemble immobilier comportant des logements faisant l'objet d'un BRS et réalisés par un bailleur social. L'adoption de cet amendement permettrait de confier la qualité de maître d'ouvrage aux bailleurs sociaux qui construisent des logements ou réhabilitent des constructions existantes dans le cadre d'un BRS.

Aujourd'hui, les organismes d'HLM peuvent déjà décider d'appliquer volontairement les règles de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique à la partie BRS d'une telle opération.

du Gouvernement ? L'article 14 de la loi de finances pour 2021 a déjà aménagé le régime d'exonération des plus-values immobilières en faveur du logement social. Cette réforme a rendu l'exonération plus efficiente, en adéquation avec son objectif de construction de logement locatif social ; elle a étendu son bénéfice aux logements construits dans le cadre d'un BRS. Je comprends l'objectif de votre amendement,

se révèle cependant d'une grande importance. Les organismes de foncier solidaire et le bail réel solidaire rendent possibles une forme d'accession à la propriété sécurisée et durablement maîtrisée qui repose sur la dissociation du foncier et du bâti, ainsi que sur le caractère reconductible du bail à chaque vente. Cela promeut le développement d'une nouvelle forme de propriété non spéculative. Opérationnels depuis 2017, les OFS connaissent un intérêt grandissant, avec 52 organismes agréés en France à ce jour. D'ici à 2024,

ailleurs, notre amendement vise à permettre de déléguer le droit de préemption urbain à un organisme de logement social pour d'autres motifs que ceux qui sont prévus, trop limitativement, à l'article L.

qui subissent une forte pression touristique et, partant, un déséquilibre social très important. L'amendement que je défends ici est issu d'une proposition de loi que vous connaissez, adoptée à l'unanimité par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

aurait abordé ce sujet. N'importe quel élu local vous dira que s'il y a un domaine où il rencontre des difficultés au quotidien, où il aimerait pouvoir mener ses projets plus simplement, c'est bien l'urbanisme. Je veux vous en donner un exemple en me faisant le porte-parole de la communauté de communes du Haut Allier, en Lozère, de ses élus et de son président, Francis Chabalier. Voilà près de six ans qu'ils se trouvent face à un mur : une double application des lois Littoral et Montagne vient réduire à néant tout projet de développement de leur territoire.

Le présent amendement, déposé par notre collègue Dany Wattebled, vise à permettre aux opérations d'aménagement de déroger à la servitude de mixité sociale lorsqu'il est justifié de l'impossibilité pour les organismes d'HLM d'y donner suite.

suppression, à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, de la condition de contiguïté des unités foncières visées par un permis d'aménager. Quel est l'avis de la commission

présent amendement de coordination juridique.

Ce dispositif, déjà ouvert dans le cadre d'une ORT, n'est pas encore utilisé à la hauteur de son potentiel. Ce faible recours s'explique en partie par la rédaction ambiguë de la loi, laquelle semble impliquer une révision préalable du plan local d'urbanisme. Un tel formalisme ne se justifie pas, dès lors que les opérations pouvant bénéficier de cette dérogation sont déjà limitées à celles spécifiquement visées par la convention de PPA. Le présent amendement vise à préciser que l'adoption des orientations

les permis d'aménager, en supprimant complètement la condition de contiguïté des unités foncières. Or l'expérimentation que nous avions votée dans la loi ÉLAN n'est pas encore arrivée à son terme et le dispositif n'a pas été évalué. Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, de le généraliser.

du code de l'environnement, en intégrant dans son dernier alinéa un droit d'option permettant au maître d'ouvrage, en accord avec l'autorité compétente, de choisir de mettre en oeuvre une seule concertation préalable- celle au titre du code de l'environnement -lorsque son projet est soumis, à la fois, à la concertation obligatoire au titre du code de l'urbanisme et aux dispositions relatives à la concertation du code de l'environnement. L'amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant dans ce droit d'option les mises en compatibilité des documents d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'un projet. L'objectif est de simplifier la mise en oeuvre de la concertation préalable pour le porteur de projet, en accord avec l'autorité compétente en matière d'urbanisme. À titre d'exemple, une opération d'infrastructure routière se trouvant en zone naturelle et urbanisée relève de deux procédures issues de deux codes : celui de l'environnement pour la partie route hors zone urbanisée, et celui de l'urbanisme pour la section située en zone urbanisée. En outre, le projet peut requérir la mise en compatibilité de documents d'urbanisme, qui, si elle est soumise à évaluation environnementale, nécessite également une concertation au titre du code de l'urbanisme. Dans un souci de lisibilité, le présent amendement vise donc à permettre au maître d'ouvrage de mettre en place pour l'ensemble de son projet et les mises en compatibilité nécessaires, avec l'accord de l'autorité compétente, la concertation préalable prévue par le code de l'environnement. Cet amendement vise par ailleurs à tenir compte dans le code de l'environnement de l'ajout, dans le cadre de la loi ASAP, d'un article 104-2-1 du code de l'urbanisme, relatif à l'évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles structurantes. Quel est l'avis de la commission

donné. Nous ne souhaitons pas revenir, huit mois après, sur des mesures adoptées dans le cadre de la loi ASAP. Il faut d'abord, me semble-t-il, mesurer l'efficacité de ces dispositions avant de les

dont les conséquences sont, de fait, beaucoup plus importantes. Nous pensons qu'il est utile de préserver, dans un document structurant tel que le PLU, les garanties en matière de concertation prévues

est à Mme Cécile Cukierman. Depuis le 1 juillet dernier, les communes ont dû, sauf mise en oeuvre de la minorité de blocage, transférer aux intercommunalités leur compétence en matière de documents d'urbanisme.

l'échelon territorial de proximité au plus près des citoyens. D'autre part, les PLU ne sont pas qu'un simple document technique d'urbanisme, mais avant tout la traduction du projet politique d'une majorité municipale élue. Aussi, imposer aux élus municipaux un PLU à la définition duquel ils n'auront pas participé et qu'ils

en indiquant que ce n'est pas aux communes de délibérer pour empêcher le transfert de compétence, mais que ce transfert est conditionné à une délibération. Nous d'autre part, d'éviter que la modification du projet d'aménagement et de développement durable n'entraîne une procédure de PLUi couvrant l'intégralité du territoire

La position constante de notre commission, depuis 2014, a été d'apporter les souplesses là où elles sont nécessaires pour appliquer les mesures de la loi ALUR, mais de ne pas revenir sur les transferts déjà réalisés. L'échelle intercommunale nous semble offrir de véritables atouts en termes de coordination de l'action des élus d'un territoire. Pour autant, nous entendons bien les demandes de nos collègues élus locaux, en particulier dans les zones rurales, qui ne souhaitent pas se voir imposer « à l'usure » un transfert de compétence auquel les communes n'auraient pas consenti

n° 1 rectifié vise à supprimer la clause de revoyure qui prévoit qu'à chaque renouvellement des équipes municipales, les communes doivent s'opposer par délibération au transfert de la compétence à l'intercommunalité si elles ne le souhaitent pas. à supprimer la disposition selon laquelle un EPCI nouvellement compétent en matière de PLU doit automatiquement élaborer un PLUi si l'un des documents communaux est révisé. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat

Ensuite, le PLUi constitue un levier pour construire et se développer. Plus de 10 000 communes en France en sont restées au règlement national d'urbanisme (RNU), qui limite fortement les droits à construire puisqu'il n'est possible de construire que dans les parties urbanisées de la commune.

Bien entendu, l'actuel dispositif de transfert ne peut pas se faire contre les élus locaux. Je rappelle qu'il existe une minorité de blocage à un seuil très bas

qui permettent des évolutions substantielles des droits à construire. D'ailleurs, projet par projet, il est possible de faire évoluer des droits à construire grâce aux déclarations de projet (DP), outils opérationnels simples que les collectivités se

Je rends hommage aux atténuations apportées à cette automaticité, que vient de nous rappeler exhaustivement Mme la ministre. Pour autant, j'ai le sentiment qu'en

Une telle diminution devra donc passer par une révision du PLU et non plus par une simple modification. Quel

les hommes et les femmes de ces territoires qui font la différence et qu'il est difficile d'avoir une vue générale pour tout l'Hexagone. Je ne dis pas que nous menons un combat d'arrière-garde, mais il faut savoir que plus de la moitié des communes

moi des mariages forcés ou contraints. Des élus qui ont connu des baisses de dotations considérables à une époque que vous connaissez bien ont couru après une échelle plus grande

et le Grand Paris, de nouvelles règles d'appréciation pour les droits à construire s'agissant des externalités positives des projets. Aujourd'hui, le respect du règlement du PLU

d'autoriser l'appréciation mutualisée, sur une surface plus grande, des externalités positives des projets de construction. Un projet qualitatif qui dépasserait les objectifs fixés en la matière se verrait attribuer une cotation qui pourrait être transférée et bénéficier à un autre projet situé sur une autre parcelle de la commune ou de l'intercommunalité,

tout en respectant les spécificités qui concernent chaque parcelle et chaque projet.

outre, les PLU, le règlement et la loi fixent déjà les règles selon lesquelles les permis seront instruits. Je ne vois pas à quel objectif supplémentaire

Vous proposez d'établir une cotation des projets assortie de certificats attestant de l'atteinte des objectifs à l'occasion des autorisations d'urbanisme. certificats pourraient être produits dans le dossier de permis de construire d'un autre projet moins bien noté pour que celui-ci soit autorisé.

précédemment, vise à soutenir l'activité touristique en zones de montagne, en apportant une réponse à la diminution progressive du nombre de logements mis en location saisonnière. C'est un véritable fléau dans nos zones de montagne depuis des années. Dans de nombreux cas, cette disparition est due à la vente du logement à un particulier qui ne le mettra plus en location. Bien entendu, la crise de la covid et la crise économique dans les stations de montagne n'ont fait qu'aggraver les choses.

Dans le cadre du plan Avenir montagnes annoncé par le Premier ministre le 27 mai, nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire l'Association nationale des maires des stations de montagne l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Syndicat national des résidences de tourisme, la Fédération des entreprises publiques locales et Domaines skiables de France. concertation avec eux, nous proposons cet amendement, qui vise à céder le droit de propriété des gestionnaires de résidences à des opérateurs fonciers chargés d'acheter des biens vendus pour les remettre en location en passant par le gestionnaire.

Cela permettra de lutter contre un autre fléau : la déqualification des résidences. Bien entendu, cela doit être étroitement encadré pour éviter tout risque de dérive.

d'autre part, des acteurs privés agréés par l'État. Nous avons souhaité encadrer très étroitement l'agrément pour vérifier l'intérêt général de la structure et prévenir les risques de collusion entre la foncière et les autres acteurs de la montagne, en particulier les gestionnaires. Cela permettra à des commerçants ou des hôteliers de la station de monter de petites structures locales. La procédure d'agrément devra associer des élus locaux, à travers la commission d'agrément qui sera mise en place. Je vous propose donc d'adopter cet amendement, qui, encore une fois, a véritablement été négocié avec tous les acteurs de la montagne.

est un enjeu important pour conserver la vitalité économique et l'attractivité de ces territoires. La multiplication des résidences secondaires- tous ceux qui habitent à proximité de stations de sports d'hiver le savent bien -est souvent vécue difficilement par les territoires concernés. Cependant, à ce stade,

pour qu'il puisse accéder à la propriété du local qui est son gagne-pain. Ouvrir une brèche dans ce principe, c'est-à-dire une possibilité de délégation de ce droit, entraînerait, me semble-t-il, un dévoiement du dispositif. On peut craindre que cela n'ouvre la porte à des pressions sur les exploitants historiques de ces hébergements pour les faire renoncer à leurs droits et les céder. outre, la finalité même du droit de priorité délégué n'est pas clairement définie. La rédaction prévue ne mentionne pas de finalité d'intérêt général, par exemple pour bénéficier du droit. La durée de l'engagement à maintenir l'activité de la résidence est de neuf ans seulement, ce qui me paraît très faible au regard de la dérogation ainsi consentie.

commerciaux à but lucratif de bénéficier de quasi-prérogatives d'ordre public, d'ordinaire réservées à la commune ou à l'EPCI, pour acquérir en priorité de tels biens. Je crains que cela ne crée d'énormes foncières privées d'acquérir peu à peu la propriété de toutes les résidences de tourisme à la ronde, et ce potentiellement au détriment de l'écosystème touristique local. À ce stade, rien ne nous garantit qu'il n'y ait pas d'opérateurs privés complètement étrangers au territoire sur lequel ils voudront récupérer ces propriétés. Nous pourrions ainsi voir des opérateurs alsaciens- je n'ai rien contre eux -venir tout récupérer en Savoie ou en Haute-Savoie. Ce serait, je le crois, de nature à porter atteinte à l'écosystème touristique local.

en introduisant une dimension départementale. Dans les faits, ces commissions ne comptent pas nécessairement de membres titulaires d'un mandat électif ou de représentants d'associations ou de fondations issus du département où se trouve le projet pour lequel un recours a été formulé. La composition de ces commissions

ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées ». Une telle situation d'éloignement des territoires, accrue par la refonte de la carte régionale, est source de difficultés dans les relations entre les élus locaux et les unités départementales de l'architecture de l'architecture et du patrimoine (UDAP). Cet amendement tend donc à prévoir que la commission est composée d'au moins un élu local ou national par département de la région et des représentants départementaux d'associations ou de fondations. Quel est l'avis de la commission des affaires

permette de travailler efficacement et dans la proximité. Cela aurait plutôt tendance à diluer encore la représentation de certains territoires en affaiblissant considérablement la part des élus. Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Nous privilégions plutôt l'aspect opérationnel.

par les arguments de Mme la rapporteure

Cet amendement vise à étendre la possibilité d'acquérir des biens sans maître au bout de dix ans, et non de trente ans, aux zones de revitalisation rurale (ZRR) et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.

d'une politique d'intérêt général pour rester conforme au droit de propriété. Ainsi, il n'est pas souhaitable de généraliser le délai de dix ans

14 900 communes ont un très grand besoin de revitalisation. La requalification du bâti existant est un levier majeur pour assurer le développement économique, en limitant l'artificialisation des sols. Tout ce qui peut y contribuer est d'intérêt général. L'enjeu est le même dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je précise que les analyses se poursuivent pour éviter toute inconstitutionnalité. Il n'est pas exclu que nous devions préciser davantage

Toutefois, les désagréments et les risques liés au mauvais entretien d'un terrain sont les mêmes qu'il s'agisse d'une parcelle bâtie ou non bâtie. Il conviendrait donc que cette disposition puisse également s'appliquer aux terrains sur lesquels se trouve un immeuble.

du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit le principe du versement d'une avance sur indemnité d'expropriation ou d'éviction, due au propriétaire ou au locataire affecté par l'opération, dès lors que les parties n'ont pu s'accorder sur le montant de l'indemnisation et que la juridiction de l'expropriation est saisie pour le fixer. L'objectif de cette mesure est de faciliter la réinstallation des personnes dans de nouveaux locaux, afin de limiter l'aggravation de leurs préjudices.

Cette inégalité a motivé la censure de l'article par le Conseil constitutionnel et son abrogation à compter du 1 mars 2022. En conséquence, afin de respecter les principes constitutionnels et de s'assurer que chaque locataire est en mesure de retrouver au plus vite et dans les meilleures conditions un nouveau logement ou un nouveau local commercial, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Celle-ci permettrait d'étendre à tous les locataires la possibilité d'obtenir un acompte, peu importe que le transfert de propriété du bien qu'ils louent ait eu lieu en vertu d'une cession amiable ou d'une ordonnance d'expropriation.

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à adapter les règles d'occupation du domaine public dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

dans le cadre des enceintes sportives dédiées aux jeux. Il est donc proposé que, dans ce cadre, les maires aient la compétence pour délivrer de plein droit ces titres d'occupation du domaine public, sans devoir

M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement concerne la procédure d'acquisition des biens sans maître. Lorsqu'un maire veut mettre en oeuvre cette procédure, qui est prévue par l'article L.

Mme la ministre. et qu'il n'encadre pas suffisamment la liste des données qui pourraient être communiquées, ce qui présente un réel risque d'inconstitutionnalité.

Il tend à prévoir que la délibération concernant la vente d'un chemin rural est dispensée d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ce chemin.

l'aliénation n'est possible que si le chemin n'est plus affecté à l'usage du public : c'est ce que doit montrer cette enquête. L'avis est donc défavorable.

permet au département d'apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l'habitat. Nous pensons que cette logique d'alliance des territoires gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu'elles appartiennent à un même pôle métropolitain. C'est un amendement de bon sens.

Par ailleurs, la couverture technique est inégale selon les territoires. Selon nous, les intercommunalités sont le niveau pertinent de la structuration de l'offre d'ingénierie publique locale. L'article 29 permet au département d'apporter un appui en ingénierie et et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l'habitat. Dans une logique d'alliance des territoires et d'ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu'elles appartiennent au même pôle métropolitain. C'est pourquoi nous proposons que toute intercommunalité membre d'un pôle métropolitain- il en existe aujourd'hui vingt-neuf sur le territoire national, d'une grande diversité et pas toujours constitués autour d'une métropole -puisse aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public en lui apportant une assistance technique adaptée pour l'élaboration du programme local de l'habitat.

Au sein du groupe RDPI, nous avons réalisé plusieurs auditions qui nous ont amenés à proposer plusieurs pistes d'amélioration. Malheureusement, plusieurs de ces amendements ont été jugés irrecevables. Je pense notamment à celui qui prévoyait l'obligation de réaliser des projets territoriaux de santé, ainsi qu'à celui qui visait à imposer la prise en compte des conseils locaux de santé mentale (CLSM) dans l'élaboration des projets territoriaux de santé. Or, dans le cadre de la santé mentale, le besoin d'une meilleure coordination et d'une meilleure collaboration a été mentionné par de nombreux acteurs auditionnés. Il nous semblait que les projets territoriaux de santé étaient des vecteurs pertinents pour assumer cette coopération entre les professionnels de santé d'un territoire, l'agence régionale Alors que 15 % des Français souffrent d'un état dépressif et 19 % d'un état anxieux, la santé mentale doit être une priorité. Nous nous félicitons, à cet égard, que les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie puissent se tenir en septembre. Je souhaitais également profiter de l'examen de ce texte de décentralisation pour mettre en lumière un exemple de collaboration efficace dans mon territoire, la Guadeloupe, où le conseil local de santé mentale permet un dialogue entre tous les acteurs clés du domaine. Ces Ces organisations sont essentielles et il est de notre rôle de parlementaires de nous assurer qu'elles puissent voir le jour sur tous nos territoires pour améliorer la prise en charge de chacun. La parole

nous interroger sur l'échec de toutes les stratégies menées pendant une vingtaine d'années par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs

modification de la majorité sénatoriale et du Gouvernement resteront à la marge. Les questions essentielles sont les missions confiées au conseil d'administration, le nombre de représentants des personnels, des usagers et des professionnels de santé, ainsi que leurs prérogatives. En attendant, la démocratie sanitaire demeurera une coquille vide. Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ? Le rapporteur

renforce également le poids des élus dans les territoires en leur accordant un tiers environ des voix au conseil d'administration, ce qui correspond à la part « assurance maladie » et à la part

a mis en tension tous les systèmes classiques de fonctionnement de nos ARS. Et pourtant, ces agences ont tenu bon et fait face aux vagues. Elles ont été capables d'accompagner les hôpitaux et les cliniques dans la déprogrammation des soins,

du covid. Les ARS ont aussi été capables d'accompagner les établissements dans la reprogrammation des soins, avec des priorisations, tout en continuant de gérer les affaires courantes : mener des politiques de prévention, de dépistage, des politiques curatives ; travailler en lien avec la santé environnementale. Les agents des ARS ne se sont jamais reposés depuis un an et demi. À aucun moment ils n'ont pu baisser la garde. Même quand les vagues diminuaient et que les hôpitaux se vidaient, leur mission restait prépondérante, tout aussi chargée au quotidien puisqu'il fallait que notre système de santé recommence à fonctionner normalement. Aujourd'hui, et depuis quelques mois, ces mêmes agences et ces mêmes agents

où l'on a parfois constaté un éloignement entre la direction de l'ARS et les délégations départementales. En cas de crise sanitaire, de toute façon, c'est le préfet qui est habilité à prendre la main sur les services de l'ARS, le délégué doit être en relation étroite avec les élus et l'ensemble des acteurs de santé du département. Dans plusieurs départements, cela se passe d'ailleurs plutôt bien, même en dehors des crises sanitaires. a cependant pas semblé très efficace, sur le plan opérationnel et pour la cohérence générale de la politique de santé régionale, de créer une rupture de lien hiérarchique

ou des ingénieurs spécialisés dans l'eau ou l'air. Ma prédécesseur Agnès Buzyn avait mis en place des emplois fonctionnels pour les délégués départementaux, afin de permettre le recrutement de managers polyvalents. Quand je dis que nous renforçons l'échelon départemental,

dont la culture traditionnelle n'était pas de partir du terrain et de travailler avec les élus locaux. Il faut que tout cela s'organise. Certaines ARS ont aussi procédé à une aspiration- c'est le cas dans ma région

une gouvernance des ARS et de leurs délégations départementales qui soit plus proche des besoins de santé. La parole

évident que les délégués territoriaux affectés à chaque département doivent être sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'ARS. Mais on parle aussi d'autorité fonctionnelle.

était possible d'imaginer qu'en restant sous l'autorité hiérarchique de son directeur régional, le délégué territorial pourrait être placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet en période de crise.

entre la liberté numérique et la liberté physique, qui peut être entravée à certains moments. C'est un autre sujet, qui avait été également relevé par le professeur Pittet. Je retire bien volontiers l'amendement. Ce qui était important, c'était de rappeler l'importance de l'échelon départemental.